Lors du jour, rappelle la suite de la discussion du projet de loi de finances, considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en application de l'article 49 aligne à 3 de la Constitution pour 2024. Dans la suite de la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 34, article d'équilibre. Nous allons donc examiner l'article d'équilibre et l'état 1 sur les voies et moyens. Je suis saisi du premier premier amendement du gouvernement, vous avez la parole monsieur le ministre, le 2300. Merci monsieur le président et bonjour à toutes et à tous. De l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement présente un amendement actualisant l'article d'équilibre afin de tenir compte des votes intervenus ici au Sénat. Les amendements que vous avez adoptés ont pour effet au global de dégrader le solde budgétaire de l'État de 0,9 milliards d'euros par rapport au projet de loi de finances issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Le solde budgétaire s'établit désormais à moins 145,3 milliards d'euros. Cette actualisation résulte de plusieurs mouvements, une hausse de 1,7 milliard d'euros de recettes fiscales, plus que compensée par une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1,6 milliard d'euros, une baisse des recettes des comptes de concours financiers de 780 millions d'euros et une diminution des recettes non fiscales de 214 millions d'euros. Les recettes fiscales nette augmentent de 1,7 milliard d'euros compte tenu des amendements adoptés en première partie. Les autres recettes fiscales est majorée de 3,348 3,348 milliard d'euros compte tenu notamment de l'amendement du rapporteur général qui supprime la prorogation en 2024 de la minoration des tarifs de l'assise sur l'électricité entraînant une hausse de recettes de 4,2 milliard d'euros. L'amendement n°210 du rapporteur général qui supprime la faculté de moduler à la hausse par arrêté les tarifs de l'assis sur le gaz naturel de façon encadrée, minorant ainsi les recettes de 1,9 milliard d'euros. D'autres amendements. Augmente la fiscalité. La hausse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 400 millions d'euros. La création d'une taxe sur les rachats d'actions, 400 millions d'euros. Le maintien à 90% du taux de la contribution sur les rentes inframarginales, 400 millions d'euros. Les recettes nettes de TICPE. pour le budget général de l'Etat sont dégradés de 987 millions d'euros du fait notamment de l'amendement 286 du sénateur Lurel qui affecte une fraction de TICPE aux collectivités et établissements publics publics territoriaux ayant adopté un plan climat-énergie entraînant une baisse de recette de l'Etat pour 1 milliard d'euros. Les recettes de TVA sont minorées de 193 millions d'euros compte tenu de l'amendement 1077 des Républicains visant à diminuer le taux de TVA sur les services de transports collectifs de voyageurs. 500 millions d'euros de recettes compensés pour partie par l'impact des amendements 245 et 246 du rapporteur général qui diminue la TVA affectée à l'audiovisuel, publique et à la sécurité sociale. Les recettes nettes d'impôts sur le revenu sont minorées de 320 millions d'euros, compte tenu notamment des amendements 321 du groupe union-centriste qui transforme en crédit d'impôts la réduction d'impôts dont bénéficient les personnes en autonomie en établissement pour une perte de recettes de 640 millions d'euros. L'amendement 1606 qui soumet a l'hier les produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie entraînant une hausse des recettes de 542 millions d'euros. L'amendement union centriste 16.05 qui soumets à l'hier les intérêts et primes dans le cadre de l'épargne de logements entraînant une hausse des recettes de 445 millions d'euros. Les recettes nettes d'impôts sur les sociétés sont minorées de 143 millions d'euros, notamment compte tenu des nouvelles informations disponibles en coordination avec le PLFSS. Enfin, les recettes non fiscales sont diminuées de 214 millions d'euros, compte tenu principalement de l'amendement du rapporteur général 236, qui affecte aux autorités organisatrices de la mobilité 250 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, la dégradation du sol budgétaire de l'État résulte du rehaussement des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales à 1,6 milliard d'euros. compte tenu de l'amendement numéro 755 du groupe union centriste qui augmente le PSR au profit encore du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 750 millions d'euros, l'amendement 618 du sénateur HENO qui crée un nouveau PSR filet de sécurité énergie pour 400 millions d'euros, l'amendement numéro 226 du rapporteur général qui relève la DGF de 170 millions d'euros, Je vais terminer. Ce n'est pas terminé. L'amendement 2280 du rapporteur général qui institue une dotation de soutien au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d'événements climatiques pour 100 millions d'euros. L'amendement L'amendement du rapporteur général qui vise à instituer une dotation de soutien exceptionnel au profit des départements confronté à une forte dégradation pour 100 millions d'euros. Quel succès monsieur le rapporteur général. Je ne peux pas en dire autant hélas. Les recettes des camps spéciaux. sont enfin minorés de 780 millions d'euros en raison de la décision de la Grèce de réaliser un remboursement par anticipation en 2023 et du fait de l'amendement du rapporteur général diminuant le montant de la TVA affectée à l'audiovisuel public. Pardonnez-moi, c'est un peu long, j'en ai terminé. En résumé, cet amendement récapitule et retrace à l'article d'équilibre les votes intervenus au Sénat au cours de la première partie du PLF. Il s'agit donc, monsieur le rapporteur général, d'un amendement technique qui traduit les votes de la majorité sénatoriale. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, vous pouvez nous présenter votre sous-amendement 2301 s'il vous plaît ? Oui Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous venez dégrainer ce que vous appelez un amendement technique. J'égrainerai moins, s'agissant d'un sous-amendement dont vous allez voir qu'il est un peu différemment de ce que vous le qualifiez donc de technique. Simplement pour préciser, nous avons terminé hier soir l'examen de la première partie du projet de loi de finances qui concerne les recettes. Effectivement, le gouvernement vient par la voix du ministre de présenter son amendement 1003 ans qui actualise l'ensemble des recettes que les votes du Sénat ont fait évoluer. Chaque mouvement fiscal hausse ou baisse d'impôts en recette en 2024 est bien pris en compte. Une première remarque, Monsieur le Ministre, le gouvernement, je viens de le constater, ne se contente pas du tout de prendre en compte les seuls votes du Sénat. En effet, Il actualise, c'est ce que vous venez de faire, des prévisions de recette de manière totalement totalement indépendante de nos votes et sans aucune justification précise. Il résulte de ces mouvements indépendants de nos votes, et vous venez de les évoquer, notamment le remboursement anticipé de la Grèce, une dégradation du solde de 1,1 milliard d'euros par rapport au texte qui nous a été transmis. 500 millions de recettes fiscales en moins sans justification précise, c'est l'évolution des recettes et je viens de le dire, 570 millions d'euros de moins que prévu parce que la Grèce nous a remboursé dès 2023 et non en 2024 un emprunt à hauteur de ce montant qui a d'ailleurs fait l'objet du contenu du projet de loi de finances de fin de gestion de l'année 2023. L'amendement que nous présente le gouvernement présente donc une dégradation du solde budgétaire de 900 millions d'euros. Mais si on enlève ces évolutions, qui ne résultent donc pas des votes du Sénat, c'est en réalité un solde amélioré de 0,2 milliards d'euros, plus de 100 millions d'euros par rapport à la copie que nous avons reçue qui sort de notre assemblée. Mais surtout, Mais surtout, Monsieur le Ministre, au-delà de quelques querelles d'évaluation de mesures sur lesquelles nous pourrons revenir, la Commission des Finances a un problème avec un des éléments que vous proposez à l'article d'équilibre et c'est l'objet du sous-amendement qu'elle a voté. En effet, vous chiffrez à 1 900 millions d'euros la perte de recette qui résulterait de l'amendement adopté par le Sénat à l'article 11 dont je vous rappelle qu'il vise à supprimer la faculté de moduler à la hausse par arrêter les tarifs de l'assise sur le gaz naturel. Cette perte de recette est en réalité nulle, car le relèvement du tarif du gaz n'est qu'une faculté accordée par la loi au gouvernement, et en outre, et en outre, Le tableau de l'évaluation préalable de l'article 11 du projet de loi de finances qu'a fourni le gouvernement et que j'ai sous les yeux ici monsieur le ministre, il est à la page 220 des évaluations préalables, et bien ce tableau il indiquait que cette mesure n'avait aucun impact en 2024. Comment donc sa suppression peut-elle aujourd'hui être chiffrée à 1900 millions d'euros ? En fait, en affichant cette perte de recette de 1900 millions d'euros, je crois simplement que vous nous révélez à cet instant votre volonté d'utiliser au maximum le levier fiscal offert par l'article 11 du PLF, en contradiction avec les chiffrages présentés lors du dépôt du texte. D'ailleurs, La Commission des Finances avait explicitement proposé la suppression de cette faculté de hausse et tarifs du gaz pour ne pas vous laisser les mains libres afin de procéder à d'éventuelles hausses massives d'impôts. Je vais citer d'ailleurs le rapport de la Commission à l'article 11 qui disait En termes de recettes budgétaires et sur le prix pour les personnes consommant le gaz, qui sont trop importantes pour que le Parlement puisse donner un blanc sang au gouvernement, l'adaptation de la mesure aux dernières prévisions d'inflation ne justifie pas que les législateurs doivent se satisfaire d'une fourchette située entre zéro et et 1,9 milliard d'euros laissés à l'appréciation du pouvoir exécutif. Il est indispensable que le gouvernement énonce clairement le tarif qu'il souhaite retenir. je regrette qu'il ait fallu attendre votre amendement à l'article d'équilibre pour apprendre en fait que vous comptiez doubler les impôts sur le gaz. Et à cet instant, je conteste vigoureusement votre amendement sur ce point et c'est absolument l'objet du sous-annement de la Commission. On ne peut pas considérer qu'un milliard neuf cent millions d'euros de recettes d'assises sur le gaz étaient intégrées au PLF puisque, je le redis, vos estimations initiales inscrites dans le document présentaient des recettes nulles. Ainsi, au total, En ne prenant en compte que les votes du Sénat et en intégrant le sous-amendement de la Commission, le solde budgétaire de l'État est donc bien amélioré d'un peu plus de 2 milliards d'euros par les votes de notre assemblée. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, qu'est l'avis du gouvernement sur ce sous-amendement 2301, s'il vous plaît ? C'est quand même très difficile de s'exprimer après une telle ovation pour le rapporteur général quand même. Mais je vais quand même essayer. Non, on n'est pas d'accord sur tout avec le rapporteur général et hélas, je crois que j'émettrai un avis défavorable sur... Je vais tenter de vous expliquer pourquoi et peut-être essayer de vous convaincre. D'abord peut-être un premier élément avant d'arriver sur la question de la fiscalité du gaz. Il y a aussi dans cet amendement que je qualifie technique, c'est normal, on actualise en fonction des événements qui se sont passés, entre l'examen à l'Assemblée nationale et aujourd'hui. Il y a effectivement la décision de la Grèce de rembourser son prêt. C'est une information qu'on actualise, il n'y a pas de difficulté. Et on actualise aussi les révisions de recettes, ce qui est toujours classique et je ne pense pas qu'il y ait là de difficultés particulières. Je pense qu'à chaque fois que vous examinez un PLF, ce type d'amendement a lieu. Je voudrais expliquer pourquoi j'ai un désaccord avec le rapporteur général sur son sous-amendement. Par ce sous-amendement, vous n'acceptez pas, j'allais dire, pour être très clair, que nous comptabilisions une perte de recette à hauteur de 1,9 milliard d'euros. Puisque l'amendement que vous avez fait voter supprime pour le gouvernement toute possibilité de relever le tarif d'assis sur le gaz. Comme il n'y a pas de possibilité d'augmenter le tarif d'assis sur le gaz, il n'y a pas de possibilité d'avoir une recette associée, donc on annule la recette associée à la hausse tarif d'assis. Je redis par ailleurs ce que j'ai dit lundi au banc, ici même. Comme nous l'avons annoncé au moment de la présentation du projet de loi de finances avec Bruno Le Maire, nous souhaitons nous saisir de la possibilité d'augmenter le tarif de l'Assis sur le gaz. le gaz. Je vous confirme que d'ici la fin de l'année, le gouvernement souhaite pouvoir réajuster à la OSS la TICGN pour remettre de la cohérence et de la clarté dans la fiscalité et dans les tarifs du gaz, sauf retournement majeur du marché. Ce qui est important. Donc la possibilité, il y a deux problèmes dans la suppression de l'amendement que vous avez voté plus tôt dans les débats, c'est qu'on a besoin de flexibilité sur ce sujet-là. Laisser cette compétence aux seuls législateurs, ça nous empêche d'ajuster en fonction de l'évolution du prix du gaz l'assise qui pèse sur le gaz. Si le prix du gaz augmente très fortement, comment le baisser ? Par voie d'arrêter, vous pouvez ajuster la fiscalité qui s'applique sur le gaz et on sait qu'on est dans une période où on a besoin de réactivité face aux évolutions de la crise. nous avons prévu à l'état B. la ligne de recette 1799 de l'état B a retenu une prévision de recette pour 2024, Monsieur le rapporteur général, à hauteur de 3,3 milliards d'euros, contre 1 milliard d'euros en 2023. Et donc dans ces 3,3 milliards d'euros, il y a bien notre estimation de 1,9 milliard d'euros qui traduit tout simplement la disposition du texte qui nous permet de prendre par arrêter une évolution des tarifs d'assises. Sur le gaz. Voilà la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs, je considère qu'effectivement il nous faut actualiser l'article d'équilibre pour tenir compte de la suppression de 1,9 milliard d'euros de recettes. Merci formellement. Oui, monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Et vous me donnerez votre avis formel sur l'amendement du gouvernement, le 2300, s'il vous plaît. Oui, monsieur le ministre, vous savez qu'en général, j'essaie de tenir l'échange de manière objective. Vous nous dites autorisation à le faire. j'ai envie de dire pourquoi pas nous on vous a dit il faut passer par le parlement ça relève des droits du parlement et on y est attaché mais j'ai envie de dire on fait bien d'y être attaché parce que vous dites donc on l'a dans un autre état c'est quand même dommage de pas remplir les cases parce que alors vous nous mettez des cases vierges sur votre document d'évaluation préalable, 24, 25, 26, 27. Et puis, je vais lire, il y a juste deux lignes en dessous du tableau. Le présent chiffrage porte sur l'utilisation de l'intégralité de facultés de majoration du taux normal d'assises sur les gaz naturels, alors 8 € du MW, dès le 1er janvier 2024. Et il est marqué en dessous le rendement associé à une majoration du tarif normal d'Assise de 1 euro s'élève à s'élève à 237,5 millions d'euros. Vous voyez, je viens de faire moi-même l'erreur. Si vous aviez été réellement transparent, vous auriez mis le conditionnel, puisque votre tableau est vierge. J'ai comme l'idée que vous avez utilisé l'ardoise magique, vous savez, on inscrit, puis finalement on se dit, il ne faut peut-être pas l'inscrire. à ce moment-là, on efface et on corrige pas le texte qui est en dessous. C'est dommage parce que finalement, dans votre volonté de transparence, vous choisissez pour décréter un milliard neuf, enfin choisir d'augmenter d'un milliard neuf mais sans le dire, vous choisissez le taux maximum. Mais dans ce cas-là, vous le dites en toute transparence et vous assumez le choix de cette augmentation de taxes. Vous nous avez dit à de multiples reprises ne pas être favorable à des hausses de taxes, Là, finalement, vous l'avez fait. Vous essayez de la faire en catémini parce que c'est vrai que quand on va gratter le contenu des taxes et assises, on ne s'y retrouve pas forcément facilement. En tous les cas, pour l'usager consommateur, il l'eût été préférable de le dire. Voilà. Donc sur l'article d'équilibre, ces remarques étant faites, monsieur le Président, je donne un avis de sagesse puisque l'objectif de toute façon, et de poursuivre la discussion. Donc on fait part de notre mécontentement et du désaccord sur une des données, notamment le fait qu'elle a été masquée, mais je souhaite en même temps que l'on poursuive pour arriver sur l'examen de la deuxième partie. Merci Monsieur le Ministre. Pas d'observation sur la concordance des temps. C'est bon. Je vais mettre donc au voie le sous-amendement. Monsieur Savoldelli, vous avez la parole. Sur le sous-amendement, monsieur Savoldelli. Monsieur le Président, vous avez raison, faut me borner un peu, moi. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, c'est pas notre groupe qui va arbitrer les chicaneries entre le gouvernement et puis la majorité sénatoriale sur les 4,4 milliards. Parce que quand même la principale recette de cette suppression des tarifs d'assises sur le gaz naturel, le volet fiscal tarifaire rapporterait artificiellement 4,4 milliards, monsieur le rapporteur général. Et moi je vous fais confiance, parce que j'ai bien regardé votre amendement, le 209, il annonce qu'il déposera des amendements de dépenses probablement pour accroître le chèque énergie. Donc voyez, comme on dit, il faut enlever la poussière sous le tapis pour avoir des moments vérités. Donc en gros, on n'aura pas un gain de 4,4 milliards, on aura peut-être, peut-être, et on verra en seconde partie ce qu'on décidera ici, on aura sans la fin du bouclier tarifaire, un surplus de 2 millions, 2 milliards de déficit supplémentaire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai une question pour le rapporteur général, pour le ministre. C'est l'évaluation du montant de la recette sur les rachats d'actions. Il est signifié là à 400 millions. Il nous paraît sous-évalué. Voilà, je vous livre cette réflexion. On n'a pas les moyens de tout instruire, mais il nous semble sous-évalué de ce point de vue-là. Par contre, ça satisfera sûrement le banc de mes amis d'en face. J'ai pu observer dans votre tableau, les uns et les autres, qu'il y a une baisse des recettes de l'impôt sur les sociétés de 143 millions d'euros. Et pourtant, et pourtant, ça va bien pour beaucoup de ces très grandes entreprises. Voilà, merci. Merci, il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Je vais donc mettre au voie ce sous-amendement 2301 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour, Le sous-amendement est donc adopté. Je vais maintenant mettre au voie l'amendement ainsi sous-amendé, le 2301 avec un avis de sagesse de la Commission qui est pour, qui est contre, il est adopté. Oui, monsieur le ministre, la parole. Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir une suspension de séance ? 5 minutes. Est-ce que, monsieur le ministre, je peux mettre au vote l'article 34 ? Sauf si c'est vraiment une demande soudaine, non, 34 ? Bon, je mets au vote l'article 34 qui est pour qui est contre. Il est adopté, monsieur le ministre. On prend cinq minutes, monsieur le ministre ? Cinq minutes. La séance est suspendue pour cinq minutes.

Je vous propose de reprendre. La séance est reprise. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. C'est pour la demande de seconde délibération que vous avez la parole. Merci Merci Monsieur le Président. En seconde, Délibération, nous présentons un nouvel amendement qui propose d'actualiser l'article liminaire à les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2024 concernant le déficit public et les grands agrégats de finances publiques compte tenu des amendements adoptés en première partie au Sénat. Pour 2024, la prévision de soldes publics s'établierait à 4,3% du PIB. Cet effet s'explique en particulier par des recettes supplémentaires induisant une augmentation du taux de prélèvement obligatoire de 44,1% à 44,3%. Cela résulte notamment de la suppression de la prorogation en 2024 de la minoration des tarifs de l'ACI sur l'électricité, entraînant une hausse de la fiscalité de plus de 4 milliards d'euros, 4,2 milliards d'euros précisément. Le solde des administrations publiques locales s'améliore notamment en raison de l'augmentation de 1,6 milliard d'euros des prélèvements sur recette au profit des collectivités territoriales et de l'affectation d'une fraction du produit de la TICPE aux collectivités territoriales pour 1 milliard d'euros. Merci monsieur le ministre. Donc j'enregistre bien votre demande officielle de seconde délibération à laquelle je réponds. En application de l'article 47 bis à lignée 1.1 du règlement, le gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article liminaire, elle est de droit. Conformement à l'article 43, lignée 5 du règlement, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de s'adopter lors de la première délibération sera envoyé à la Commission, qui doit présenter un nouveau rapport. L'amendement de seconde délibération vous a été distribué, il est sur table, il est en cours de distribution. La Commission s'étant déjà réuni, nous allons procéder à la seconde délibération, Monsieur le Président. Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43 alinéa 6 du règlement dans sa seconde délibération. Le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la Commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. Monsieur le ministre, je crois que vous avez présenté votre article liminaire. Je vais donc demander l'avis de la Commission. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Ce Ce sera à nouveau un avis de sagesse au regard de la présentation qui a été faite par le ministre et en intégrant les derniers paramètres comme cela a été rappelé. Merci. Je vais donc mettre au voire cet amendement A1, à la suite de la nouvelle délibération, avec un avis de sagesse de la Commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je mets au voie maintenant l'article liminaire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Avant de passer au vote sur l'ensemble de la première partie, je vais donner la parole à ceux de notre collègue qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. Je rappelle au Sénat que conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et à l'article 47 bis à ligne A2 de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidé par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de 5 minutes pour ses explications de vote, à raison d'un orateur par groupe, l'orateur des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe disposant de 3 minutes. La parole est d'abord à madame Carrère. Je vous remercie. Tous nos remerciements d'abord au Président Claude Rénal qui n'a cessé de veiller avec une bienveillante autorité à ce que la durée de nos échanges respecte le délai constitutionnel. Je félicite aussi notre rapporteur général Jean-François Husson pour son travail, son écoute et son souci d'assurer toujours la cohérence de nos votes, sans oublier bien sûr Christine Lavarde, notre collègue, qui a vaillamment siégé au banc de la Commission dimanche dernier. Mes chers collègues, nous voterons cette première partie, mais je veux partager ici avec vous les raisons pour lesquelles cette année, le vote de notre groupe sera avant tout un vote en responsabilité. Ce sera un vote en responsabilité d'abord dans l'intérêt de la démocratie. À l'Assemblée nationale, en effet, le gouvernement a choisi d'avoir recours au 49.3 dès le début et non à l'issue des débats. Dès lors, tous les débats si nécessaires à un texte aussi essentiel que le budget de l'État n'ont eu lieu qu'au Sénat et n'auront lieu qu'au Sénat. On a même vu tout à l'heure à quel point le gouvernement aimerait même se passer du Parlement pour relever la fiscalité, ce qui était inacceptable. Il est donc de notre responsabilité d'examiner ici la deuxième partie du projet de loi de finance. Et pourtant, nous aurions pu dénoncer par notre vote les conditions si particulières de nos travaux. Car non seulement il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, mais le texte qui nous a été soumis était passé de 59 à 234 articles, soit au total trois quarts des articles du projet de loi de finances qui n'auront été examinés ni par le Conseil d'État ni par l'Assemblée. C'est tout de même une drôle de lecture de l'article 39 de la Constitution, qui dispose que les procès de loi sont délibérés par le gouvernement à préavis du Conseil d'État et d'autre part que les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Si notre vote est avant tout un vote de responsabilité, c'est aussi, il faut bien le dire, parce que dans certains cas, des majorités de circonstances ont abouti à des choix qui ne sont pas les nôtres. Je pense par exemple au rejet de la hausse du plafond du caution familiale que nous avions proposé pour le pouvoir d'achat des familles. Je pense aussi naturellement au vote d'un alourdissement de la fiscalité sur l'épargne de logements et l'assurance vie. Ils sont à rebours de notre ligne constante de ne pas augmenter la fiscalité et de préserver les classes moyennes. Tout n'a pas été négatif, bien sûr, loin sans faux. Nous félicitons notamment de l'adoption de propositions visant à répondre à la crise du logement, mais aussi en faveur des collectivités territoriales, ainsi que des entreprises s'agissant du régime de la procession. De nombreuses dispositions ont également fait l'objet d'une belle unanimité. Je pense par exemple au financement du Centre national de la musique ou à la suppression des scandaleux avantages fiscaux que vous souhaitez accorder à la FIFA. Et je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir tenir compte de l'unanimité qui s'est dégagée sur ces bancs pour que louer sur Airbnb ne soit pas fiscalement plus avantageux que l'allocation de longue durée, qu'elle soit meublée ou non. Je pense aussi aux solutions que nous avons trouvées sur les ZDR ou le PTZ, à l'adoption de notre proposition si audacieuse d'affectation de 250 millions de quotas carbone au financement des transports collectifs, à la hausse de la DGF, à celle de la DPEL et à suppression du critère de potentiel financier, ou encore à la mise en place pour les collectivités d'un mécanisme d'étalement des remboursements du filet de sécurité à inflation. Monsieur le ministre, comme vous en avez aimablement égrené la menace tout au long de notre débat avec votre compteur dont nous aurions aimé partager les données, vous nous reprochez enfin de discussion d'avoir dégradé le sol budgétaire. Eh bien non D'une part, nous n'adhérons pas à tous les chiffrages à la louche et invérifiables de nos amendements, pas plus d'ailleurs qu'au chiffrage de certains de vos propres amendements. De même que nous n'adhérions pas à vos prévisions de croissance pour 2024, que l'OCDE vient de démentir à son tour, avec malheureusement une prévision à 0,8 qui ne nous réjouit pas plus que vous. D'autre part, nous allons vous présenter plus de 5 milliards d'euros d'économies afin de permettre un retour sous les 3% dès 2025. Le gouvernement, je le rappelle, prévoit de franchir ce cap qu'en 2027, ce qui ferait de la France, à la fin du quinquennat, le pays européen ayant le déficit public le plus important. Tel n'est pas notre projet pour le pays. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera la première partie du projet de loi de finance pour 2024. Je vous remercie. Merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Jurek. Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez trois minutes, cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers collègues, Nous voilà donc réunis pour donner notre assentiment à la première partie du projet de loi de finances. Mais que voulons-nous ? De quoi débattons-nous ? Cite au sorti de ce palais, nous savons très bien que le gouvernement dégainera un énième article 49.3 dans le mépris complet des assemblées. Le ministre de l'économie, qui ne daigne même plus venir défendre son texte devant nous, est aussi bon gestionnaire que romancier. Contrairement aux belles phrases aux milliards énumérés, nous voilà donc devant un budget de faillite. Ce budget tient aussi d'un paradoxe terrible pour nos compatriotes. La pression fiscale demeure la plus élevée de l'Union européenne, si ce n'est du monde, et parallèlement, notre déficit budgétaire et notre dette continuent de croître. Les charges de la dette représenteront bientôt le premier budget de l'État devant l'éducation nationale, le pseudo parti du bon sens, les mauxards de la finance autoproclamés cumulent les mauvaises notes et continuent par ailleurs d'aggraver lourdement notre endettement. Par ailleurs, si la France est à l'euro près, où sont les nouvelles recettes ? Aucune mesure pour faire payer la richesse financière n'a été retenue par le gouvernement, aucune mesure pour davantage taxer les GAFAM et les grandes entreprises, si ce n'est un impôt européen minime, fruit des étreintes scabreuses entre l'Union européenne et le pouvoir des lobbies. L'Union Européenne, parlons-en, avec 24 milliards d'euros et une contribution nette beaucoup trop nette envoyée à Bruxelles. La France est le dindon de la farce de la construction communautaire. Certes, la dîme bruxelloise est allégée en 2024. Élections européennes obligent, mais elle ne cessera de croître dans les années à venir, alors que vous prévoyez d'étendre encore plus l'Union Européenne en y ajoutant 5 ou 6 pays. Vous nous parlez d'avenir, la belle affaire. Aucune mesure fiscale ou budgétaire ne vient soutenir notre natalité à tonne, pourtant pilier de toute prospérité. Les familles françaises, prises entre l'enclume de l'inflation et le marteau de l'impôt, n'auront droit qu'à des chèques, faibles analogiques contre la gangrène qui ronge notre pouvoir de vivre et plonge nombre de nos concitoyens dans la plus sombre des précarités. Vous nous parlez d'investissement et de transition écologique, mais vous semblez oublier que vous vous en défossez en premier lieu sur les collectivités territoriales, et pour ces dernières, le mépris se poursuit. Vous nous présentez avec tombours et trompettes une augmentation de la DGF de 200 millions, très bien, mais vous oubliez que ces 40 milliards d'impositions locales qui ont disparu des caisses des collectivités territoriales depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Solzhenitsyn disait « ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils continuent de mentir ». Au lieu de chercher la solution miracle pour battre Marine Le Pen en 2027, vous seriez plus inspiré de chercher à sauver le pays. Contre le mensonge qu'est votre optimisme, contre la faillite qu'est votre projet de loi de finances, nous votre don contre cette première partie. Je vous remercie.

Monsieur le Président, monsieur le Ministre, monsieur le Président de la Commission des Finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, Nous votons aujourd'hui un budget qui est placé sous le signe de l'inflation. Certes, la hausse des prix serait limitée l'an prochain à 2,6 %, une bonne nouvelle pour nos compatriotes. Mais je ne parle pas de cette inflation-là. Je veux parler de l'inflation législative. Nous avons, en effet, de nouveau battu notre propre record du nombre d'amendements. Une hausse de près de 40 % par rapport à l'an passé qui était déjà une année record. Plus de 2000 amendements déposés en première partie. Seule une minorité d'entre eux améliore les recettes. La majorité les dégrade. Mais au-delà de l'impact sur le solde public, c'est surtout l'impact de la lisibilité de notre droit qui s'avère fâcheux. Comment espérer redonner puissance et efficacité à l'action publique si les lois de finances ne simplifient rien et complexifient tout ? Les élus locaux, vous le savez mes chers collègues, n'en peuvent plus. Bien sûr, notre groupe a contribué à cette effusion législative. Mais en valeurs relatives comme en valeurs absolues, nous avons fait preuve de sobriété parce que nous sommes le groupe qui en a déposé le moins. Le président Larcher ne cesse de nous le répéter. Nous devons moins légiférer pour mieux légiférer. C'est une sagesse toute romaine que je partage. En matière budgétaire, nous n'avons plus de choix. Si cette inflation se poursuit, nous n'aurons pratiquement plus le temps d'examiner tous les amendements, car le calendrier budgétaire, lui, reste rigide. Hausse du nombre d'amendements d'une part, contrainte du calendrier d'autre part, Nos débats sont mécaniquement comprimés et c'est notre démocratie délibérative qui en pâtit. Les trois protagonistes de ces débats n'ont pourtant pas ménagé leur peine et je tiens à saluer leurs efforts. Notre rapporteur général qui a su résumer ses avis à l'essentiel. Notre président de commission qui a su nous rappeler à la concision. Monsieur le ministre, vous avez défendu votre premier budget également avec calme et précision. Mais malgré la vigilance de chacun, le budget sort du Sénat alourdi de nouvelles taxes, allégé de nouvelles niches. Notre fiscalité, à l'image un peu de notre tour Eiffel, devient une structure qui tient autant de l'industrie lourde que de la toile d'araignée. Dans ce budget, tout n'est pas ajouté et loin s'en faut. Plusieurs mesures votées ont un impact positif, notamment pour les collectivités. Je pense bien évidemment que cela a été rappelé par mes collègues à la réforme des ZRR via le dispositif France Rurales, qui répond à la plupart de nos revendications. Plusieurs mesures en faveur de l'innovation ont également été adoptées. Elles visent à soutenir les investissements pour nos startups et donc à préparer la richesse de demain. Je pense évidemment au crédit d'impôt innovation. Il y a plus d'un an, j'avais rapporté au nom du groupe Les Indépendants une mission d'information sur la recherche et l'innovation au service de la réindustrialisation de nos territoires. Ce dispositif avait été identifié comme décisif pour le soutien des start-up industriels qui ont, Monsieur le Ministre, vous le savez, des besoins sui generis. C'est pourquoi je vous ai proposé de proroger de deux ans ce dispositif, d'en relever le plafond des dépenses éligibles en le faisant passer à 800 000 euros. D'autres mesures visent à permettre d'accélérer la transition écologique des territoires. C'est le cas par exemple des amendements pour développer l'autoconsommation d'énergie renouvelable qui permet de décentraliser nos capacités de production pour consommer l'énergie en circuit court. ou encore le rétrophite de véhicules thermiques à l'électricité ou à l'hydrogène qui lui permet de verdir nos flottes et de contribuer à l'économie circulaire. Je ne ferai pas un embouteil à la prévère de toutes ces mesures qui sont pertinentes, mais je tiens à en mentionner deux qui n'ont malheureusement pas été retenues et concernent la préservation de notre patrimoine religieux. La première, défendue par mon excellent collègue Emmanuel Capu, visait à intégrer les églises des communes nouvelles dans la souscription nationale en faveur du patrimoine religieux, tel que voulu par le Président de la République lui-même. Il n'est pas logique qu'elles en soient exclus et j'espère que le tir pourra être rectifié d'ici à l'adoption finale du texte. La seconde concernait la reconversion du site de l'abbaye de Clairvaux. J'ai déjà eu l'occasion, Monsieur le Ministre, de vous alerter de vous alerter sur ce sujet, la rénovation de ce site exceptionnel doit devenir une priorité nationale. Aujourd'hui, les financements privés manquent sur le volet travaux et activités non lucratives, notamment culturelles. Il n'y a pas de modèle économique viable sans mécénat bonifié sur ces volets. J'espère que nous pourrons ensemble trouver rapidement une solution opérante pour ce dossier au bois de premier plan. Chers collègues, la parole est maintenant à monsieur... Oui, allez-y, allez-y. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, chers collègues. Monsieur Delcroz, vous avez la parole pour le groupe union centristes. Vous avez cinq minutes. Monsieur le Président, monsieur le Ministre, monsieur le Président de la Commission des Finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, Tout au long de cette première partie, le groupe de l'Union centriste a présenté des propositions autour d'un cap clair. Réduire le déficit budgétaire par la mise en œuvre d'une politique fiscale plus juste visant les très grosses fortunes et non les classes moyennes comme je l'ai entendu. Et nous nous réjouissons de l'absorption par le Sénat de plusieurs amendements allant dans ce sens. Le renforcement de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, elle cible particulièrement les superdividendes qui échappent à la progressivité de l'impôt depuis la mise en place du PFE en 2018. La réforme de l'Exit Tax qui garantira que les contribuables, contrôlant une société ayant bénéficié du soutien financier massif de l'État, ne puissent échapper à l'impôt sur les plus-values en se délocalisant seulement deux années à l'étranger avant de les céder. La taxation des rachats d'actions par les très grandes entreprises, une pratique qui a explosé ces dernières années. Il s'agit de les encourager à investir dans l'économie réelle plutôt qu'à faire monter le cours des actions. La suppression de plusieurs niches fiscales dans un tripoblégatif de redressement des finances publiques, d'efficacité économique et d'équité sociale. le renforcement du plan de lutte contre la fraude fiscale ou encore le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive pour une taxation plus juste des actifs financiers improductifs. Nous avons aussi défendu la mise en œuvre de politiques publiques utiles par l'adoption de plusieurs amendements, comme par exemple le maintien du prêt à taux zéro en zone rurale pour ne pas pénaliser les primo-accédents souhaités résider à la campagne. ou encore l'augmentation de la DGF, notamment pour rétablir la hausse de la DSR au niveau de 2023. Enfin, la réforme des ZRR. Je ne peux pas passer sous silence ce sujet. Si sur la forme, son examen à mon sens trop précipité a parfois conduit à un peu de confusion, sur le fond, et c'est cela qui compte au fond, le résultat est à la hauteur des enjeux grâce à une convergence quasi totale entre le Sénat et le gouvernement au seul bénéfice des territoires ruraux. Sur cette question à fort enjeu et à fort portée symbolique, je tiens à remercier particulièrement d'abord Madame la Première Ministre d'avoir inscrit la pérennisation de ce dispositif à plusieurs reprises menacées de disparition dans le plan France ruralité annoncé en juillet dernier et sa concrétisation dans la loi de finances pour 2024 sous la forme de France ruralité revétalisation. Je veux remercier aussi la ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, qui durant plusieurs mois a joué la carte de la concertation avec les parlementaires et les associations d'élus pour rechercher le consensus le plus large autour de la meilleure réforme, améliorant ainsi la copie initiale du gouvernement. Enfin, merci à vous Monsieur le Ministre présent tout au long de ce débat pour votre écoute et votre ouverture sur cette question importante. L'accord conclut entre le gouvernement et le Sénat. C'est traduit par un vote unanime ou quasi-unanime, rassemblant toutes les sensibilités et tous les territoires autour d'un projet commun. Un projet qui répond aux besoins des territoires ruraux et un message positif, encourageant, adressé au secteur rural et c'est important. Alors Monsieur le Ministre, Là, du coup, je m'adresse à vous. Après cet accord trouvé grâce à une réelle concertation, après ce vote unanime au Sénat, nous comptons sur le gouvernement pour que le texte définitif qui pourrait faire l'objet d'un 49.3 respecte l'accord trouvé avec la Chambre des territoires. Voilà un balayage rapide des rapports de notre groupe qui, au global, ça a été rappelé, contribuent au redressement des finances publiques grâce aux économies réalisées. Il ressort du Sénat, à notre sens, un texte solide qui répond aux enjeux du moment et nous le voterons. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame Ghislaine Senet pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Vous avez cinq minutes, cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Nous voilà donc arrivés au bout de ces nombreuses heures de débats sur les recettes du budget de l'État 2024, au cours desquelles nous avons examiné près de 2 400 amendements. Cette inflation des propositions sénatoriales pourrait être perçue comme un symptôme de vitalité démocratique. Or, je crains qu'elle reflète davantage les frustrations d'une représentation nationale qui se voit baillonnée au palais Bourbon. Nous aimerions, je crois tous, pouvoir partager l'examen du budget de notre nation avec nos collègues députés. Malgré l'alerte que le groupe écologiste Solidarité et territoire vous a signifié à l'ouverture de ces débats, ce budget et recette ne répond pas à l'urgence d'une action d'envergure en faveur de la transition climatique dans laquelle la France doit impérativement s'engager si elle veut assurer son avenir dans ce monde menacé par l'hyperactivité humaine et le réchauffement global. C'est en effet ce que préconisent Jean-Pizani Ferri et Selma Mahfouz dans leur fameux rapport, dont on a bien compris que vous n'aimiez pas que l'on se réfère, alors même qu'il fait, au contraire, montre d'une grande objectivité. Ce rapport chiffre à 66 milliards d'euros par an le montant des investissements nécessaires pour financer la transition et pour que la France s'aligne enfin sur la trajectoire de neutralité climatique qu'elle s'est fixée. Vous avez osé assumer que cette année vous y répondiez à hauteur de 30%, le reste étant à la charge des collectivités qui, si elles participent en effet à 70% de l'investissement public, doivent aussi assumer bien d'autres charges et compétences transférées et non compensées, mais de cela nous en reparlerons dans la seconde partie de ce budget. Revenons plutôt à la préconisation de ce rapport demandé par madame la première ministre, rappelons-le, et qui préconise deux solutions de financement, le recours à l'emprunt pour les dépenses vertes et la taxation provisoire des plus hauts patrimoines financiers. Force a été de constater tout au long de ces débats que vous ne vouliez ni de l'un ni de l'autre. Alors, nous avons tenté de corriger le tir en vous présentant des propositions de bon sens, parfois ambitieuses, mais vous les avez pour beaucoup balayées, monsieur le ministre, parfois d'un revers de la main. Nous avons tout d'abord proposé de demander à chacun de contribuer à la hauteur de ses capacités à l'effort collectif pour transformer notre société. Vous et la Commission des Finances y avez émis un avis défavorable. Nous vous avons ensuite proposé de mettre fin rapidement à l'ensemble des dépenses fiscales néfastes pour le climat dont la seule existence dans le contexte actuel d'emballement est une insulte aux générations futures et à l'avenir de notre société. Là encore, vous avez émis un avis défavorable. Nous vous avons enfin proposé d'instaurer une fiscalité favorable pour les secteurs d'avenir que constituent les transports des carbonés, les énergies renouvelables ou l'agriculture durable. Là encore, avis défavorable. Alors, quelques avancées ont tout de même été obtenies de ci de là, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour assurer la transition climatique ni pour rétablir plus de justice sociale. Et à ce propos, je voudrais tout de même saluer l'adoption de l'amendement de nos collègues centristes votés avec les voix de la gauche et des écologistes et qui visent à permettre de renforcer la fiscalité sur les hauts revenus. S'il est impératif en effet de demander aux plus aisés de participer selon leurs capacités à l'effort collectif, j'ai malheureusement bien peur que cet amendement ne passe sous les fourches codines d'un prochain 49.3 à l'Assemblée. Frêchement élue, je réalise à quel point le chemin est encore long, ici à droite de cet hémicycle, pour accepter de sortir du dogme de la rigueur budgétaire et que nous sommes bien loin de changer de braquet. Nous concernons, cela fait 40 ans que les écologistes défendent l'impérieuse nécessité d'un changement de modèle. Il n'est plus temps de tergiverser. Car on le sait désormais, le coût de l'inaction climatique sera largement plus élevé que le coût de la transition. Une étude de la Banque centrale européenne montre que clairement, à partir de plusieurs scénarios, plus on attendra pour agir, plus le coût financier sera élevé pour les entreprises et les ménages. C'est la raison pour laquelle mon groupe votera contre cette première partie du budget. Et si vous me permettez un dernier mot Monsieur le Ministre, la France a deux grandes forces sur lesquelles vous devriez vous appuyer pour réussir l'effort de transition. Tout d'abord l'administration qui aujourd'hui s'engage fortement dans la tenue des objectifs fixés. Et puis notre pays est également riche de ces 520 000 élus volontaires engagés qui sont prêts à s'investir pour transformer leur territoire et répondre aux enjeux à venir. Alors sortez de votre frilosité, tracez une ligne claire et ambitieuse, donnez surtout les moyens pour que nous puissions la réaliser collectivement et alors nous pourrions entamer avec efficacité et intelligence le tournant dont la France a tant besoin. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCOK. Vous avez 5 minutes, cher collègue. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, monsieur le Président de la Commission, monsieur le Ministre, mes chers collègues. La majorité sénatoriale votera la première partie de ce budget 2024, j'irais dire comme elle l'a fait pour le budget de la sécurité sociale. C'est une forme de continuité. Ce faisant, elle donnait son aval au rabot, je me rappelle au nom de l'efficience, de 500 millions d'euros pour les hôpitaux, en décalage total avec les 2 milliards réclamés par la fédération hospitalière de France, qui était la réponse face à l'insécurité sanitaire. Le déficit provient du refus en bloc, de prélever sur le capital le financement des besoins de santé publique et ce projet de loi de finances s'inscrit dans la même logique. L'examen au Sénat aménage les plus riches, les patrimoines mirobolants et les revenus financiers. Exception faite d'une contribution sur les rachats d'actions des grandes entreprises. Cette mesure pour laquelle notre groupe s'est particulièrement battu et conteste le fait qu'elle soit évaluée seulement à 400 millions d'euros. Mais on verra la suite. Les propositions du groupe centriste ciblent les ménages et corrigent à la marge certaines injustices. J'irais dire, mais il y a un mai, mais c'est un mai majeur, mes chers collègues. Jamais les profits exponentiels du 4,40 sont mis à contribution. Je le rappelle, 80 milliards d'euros pour le premier semestre 2023. En gros, le capital s'en sort bien, les inégalités sociales et fiscales subsistent. La droite sanatoriale a contribué à accroître comme jamais auparavant les déficits publics. Elle a prolongé et renforcé dans ce projet de loi des niches fiscales non évaluées coûteuses. La partie recette est dévoyée et d'ailleurs elle porte mal son nom quand n'y sont votés que des dépenses en faveur des plus aisées. Au prétexte de résoudre la crise du logement, le président Retailleau et ses collègues ont fait voter un relèvement de l'abattement pour les donations pour l'acquisition d'une résidence principale à 150 000 euros. Il nous faut tenir, mes chers collègues, un discours de vérité. 87% des Français perçoivent un héritage total dans toute leur vie de moins de 100 000 euros. Donc ce rehaussement, c'est une mesure à 2 milliards au moins pour les riches. Parce que le logement, c'est un prétexte. L'État partenaire, associé aux plus riches, aux banques et aux organisations privées des marchés financiers, est le choix stratégique de la droite. Les plus modestes, le logement social est lui le grand absent de nos débats. 80% des demandes dans le parc social sont éconduites. 2,14 millions de demandes en attente qui nécessiteraient de construire 198 000 logements sociaux par an entre 2024 et 2040. En 2023, seuls 90 000 sont sortis de terre. Nous touchons le fond. Le gouvernement et la droite sénatoriale refusent de désamorcer ce qu'on appelle cette bombe à retardement. Pour les collectivités, la perte de marches financières est toujours d'actualité. Certes, des amendements défendus notamment par notre groupe renforcent la taxe sur les logements vacants. Mais pas d'indexation de la DGF sur l'inflation, marquant une baisse de 5,6 milliards, tout transfert confondu en euro-contents. poursuite de la suppression de 19,6 milliards d'euros de CVAE et la perte potentielle de la dynamique pour les communes, pas de déplafonnement ni de corrélation réelle entre la taxe foncière et la taxe sur les résidences secondaires. La centralisation des ressources des collectivités est un fait avéré. Des dotations à l'investissement encadrés par les préfets. C'est une conception de l'autonomie financière quand même très étroite. Parallèlement, les collectivités sont traitées comme des sous-traitants des politiques nationales. C'est vrai pour le service public de la petite enfance, c'est vrai pour la transition écologique et je pourrais prendre d'autres sujets. Aussi, monsieur le ministre, chers collègues aussi, la dotation de 100 millions d'euros supplémentaires pour les départements, évidemment contre l'avis du gouvernement. Mais elle s'avère totalement insuffisante. Seulement dans mon département, le Val-de-Marne, c'est déjà 90 millions d'euros probablement d'écart sur les DMTO. Qu'est-ce qui va rester pour les autres ? Alors qu'ici, tous mes collègues de toute sensibilité disent que des départements vont peut-être déposer le bilan. de tels écarts des droits de mutation. Et alors, après, passons aux entreprises et les ménages. Ils ont aussi pas tellement été aidés. Alors les ménages, non, mais les entreprises, pas tant que ça. Parce que la dette privée est un tabou. On n'a pas le droit, on n'en parle jamais ici. Mais la dette privée, c'est 162% du PIB. La dette publique a presque un côté, fait un peu pâle figure. Et nous vous conseillons d'ailleurs la lecture du livre de mon collègue Eric Bocquet qui s'appelle « La dette à perpètes ». Le tout, malgré le florilège de crédits d'impôts et autres aides en tout genre, ce n'est pas la fiscalité et les cotisations sociales qui endettent les entreprises, c'est le coût du capital. Vous comprendrez que nous ne faisons pas confiance aux 49.3 et vous avez bien compris que nous avons monté contre ce texte. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Biac pour le groupe RDSE. Vous avez 5 minutes, chers collègues.

M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur général, M. le Président de la Commission de Finances, mes chers collègues, après trois projets de loi de finances élaborés dans des contextes difficiles, dont les budgets furent marqués successivement par la crise sanitaire, les élections, je crois, et la crise énergétique, ce budget 2024 intervient dans une situation quasi normale, le PIB revenant au niveau de 2019. La partie recette du projet de loi des finances pour 2024 présente des prévisions gouvernementales plus optimistes que celles de tous les économistes, notamment en ce qui concerne la croissance. Pendant ce temps, la dette continue de croître et la hausse des taux d'intérêt va peser lourdement sur les comptes publics. Le déficit budgétaire se maintient très haut au niveau de la crise sanitaire

Je reviendrai rapidement sur mon amendement de l'article 28 où je demandais la suppression des agences de l'eau. Amendement quelque peu provocateur qui a été rejeté, je m'y attendais. Je voulais par cela engager une dynamique pour réduire les dépenses de fonctionnement des auteurs publics et des administrations centrales. Le constat est accablable. Nous avons trop d'opérateurs qui consomment en frais administratifs des crédits qui seraient plus utiles si ils étaient versés directement aux collectivités pour les services opérationnels. Comment peut-on justifier que les frais généraux, les frais administratifs soient deux fois plus élevés en France que chez nos voisins européens. Comment expliquer à nos concitoyens que nous sommes les champions du monde de déprélevements obligatoires, que les dépenses de personnel ne cessent d'augmenter, mais qu'en même temps, sur tout le territoire, il manque des enseignants, des policiers et que les déserts médicaux se multiplient Les idées locaux et les maires dénoncent tous les lourdeurs administratives. En Alcongré, le maire de Casoul-des-Bégiers, me faisait part de sa volonté de réaliser une centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge. Quatre ans, ans que l'administration lui demande étude, étude, étude, rapport, et pendant ce temps, cette centrale photovoltaïque reste dans les cartons. Les chefs d'entreprise que je rencontre, ça doit être pareil pour mon collègue. Il y en a marre de l'administration qui nous étouffe, laissez-nous faire. Quant aux agriculteurs, Eh bien, là aussi, ils disent de passer plus de temps devant leur ordinateur que sur le tracteur. Ce constat n'est certes pas nouveau. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Déjà, le président Pompidou demandait à l'administration, je cite ses propos, que ça ne me permettait pas d'arrêter d'emmerder les Français. On en est toujours là. Pour conclure cette explication de vote au nom du groupe RDSE sur le volet recette du budget 2024, je tiens à souligner quand même les avancées escrites dans le texte par le Sénat, avec 1,615 milliards d'euros supplémentaires pour les collectivités locales. Le Sénat, c'est la chambre des territoires, et nous le prouvons. Rapidement, l'abonnement du fonds d'urgence pour les inondations, et une dotation incendie pour les communes rurales, la revalorisation de 100 millions de la DGF, l'élargissement du prêt à taux zéro pour tous les territoires, la prolongation du fil de sécurité énergétique pour les collectivités, 100 millions insuffisants mais enfin pour les départements, l'élargissement de la DPL aux communes de moins de 1000 habitants sans condition de ressources et 3000 communes supplémentaires éligibles, et le FFR, en regrettant toutefois le rejet de l'amendement RDSE pour le département du Lot, ce département qui est exclu pour quelques habitants en raison d'un problème de procédure de règlement où l'amendement du RDSE est tombé. Je n'oublierai pas les dotations confortées pour les chambres consulaires, chambres de culture, chambres de commerce et industrie et chambres des métiers qui ont trouvé le soutien du Sénat. Pour conclure, je voudrais remercier monsieur le ministre, monsieur le Président, monsieur le rapporteur pour leur écoute et pour leur pédagogie. Alors, comme la majorité des membres du RDSE, je voterai cette première partie du budget 2024, tout d'abord pour les avancées qu'elle contient, mais aussi afin afin de pouvoir examiner le volet dépenses, car, vous le savez, le groupe RDSE est très attaché à la poursuite du débat parlementaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. En retrouvant mon intervention prononcée ici même l'an dernier, j'ai constaté que le nombre d'amendements déposés avait déjà dépassé tous les records. Nous en étions alors à 1741, bien loin des 2300 déposés cette année. Comme vous l'avez proposé l'an dernier, Monsieur le Président de la Commission des Finances, cher Claude Rénal, je crois que nous devons nous interroger sur cette inflation législative. Quelles en sont les causes ? Et surtout, comment la contrecarrer pour éviter de se retrouver face aux dépôts de 5 000 amendements dans trois ans. Mes chers collègues, les débats de cette première partie du budget se sont tenus dans une ambiance assez étrange et ce dès le départ lors du rejet de l'amendement déposé par Bruno Rotaillot sous le conscience familiale qui permet de vous rappeler a récouté plus de 1,5 milliard d'euros et pour les plus favorisés, suivi d'un nouveau revers pour le groupe majoritaire sur l'assurance vie. Depuis juin 2022, les oppositions à la majorité présidentielle ne cessent de pointer du doigt l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et bien, chers collègues de la majorité sédatoriale, vous venez également de faire l'expérience des charmes de la majorité relative. Et cette première partie ne ressemble en fin de compte qu'à un tissu de contradiction, entre les taxes nouvelles votées à votre corps défendant, un grand nombre de mesures nouvelles particulièrement coûteuses et des niches fiscales comme s'il en pleuvait. Par ailleurs, alors que vous ne cessez d'appeler la maîtrise des finances publiques, nous avons pu constater une fois de plus votre tendance à l'incohérence de ce discours, s'agissant des collectivités. Vous avez voté plus d'un 1,6 milliard d'euros supplémentaires. Alors oui, on est dans la chambre des territoires, mais je crois que c'est incompatible avec un discours de responsabilité, de redressement des comptes publics. Le paradoxe, c'est que vous profitez pour financer ces dépenses des recettes votées contre la ligne de votre groupe. Même le président Rotailleau est monté au créneau à un moment donné pour mettre le holà à vos dépenses excessives. Je pense à la compensation rétroactive pour les dépenses des communes sous les aménagements de terrain ou encore au filet de sécurité relatif à l'énergie. On a bien senti une gêne sur ces bancs au moment des votes. Autre contradiction, je n'ai toujours pas compris la position de la majorité sénatoriale sur la suppression progressive de la CVAE. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Sauf si vous êtes devenus adeptes en même temps. Cela étant, cette première partie du budget contient des avancées que je tiens à souligner. À commencer par la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les tensions survenues dans l'hémicycle lorsque le sujet a été abordé sont assez déconcertantes. Cette année, le ministre nous propose pour la première fois une décorrélation de cette taxe et de la taxe foncière. C'est une avancée historique. Mais notre hémicycle a été très agité à ce moment-là. Notre groupe RDPI vous est reconnaissant, monsieur le ministre, pour votre engagement sur le sujet. Notre groupe tient également à saluer l'adoption d'une partie significative de nos amendements. Sur les 18 déposés, 10 ont été adoptés. Je pense à la prolongation de la réduction du taux d'impôt pour les dons et versements effectués au profit des organismes d'aide alimentaire aux plus démunis qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur prodiguent les soins essentiels. Je pense également à nos amendements pourtant sur le logement, un secteur actuellement en crise. Il y a celui sur le pré-avance mutation destiné au ménage ressources modestes souhaitant financer des travaux de rénovation permettant d'améliorer la performance énergétique de nos logements ou encore la possibilité de souscrire un éco-pré à taux zéro complémentaire quelle que soit la nature des travaux financés par l'avance initiale et sans oublier la prorogation du dispositif de Normandie jusqu'en 2026. Je pense enfin à nos amendements adoptés relatifs aux Chambres d'Agriculture et aux Chambres de Commerce et d'Industrie dont les moyens financiers seront préservés ou renforcés. Cependant, compte tenu des amendements adoptés sous le fil des Sécurité, les dépenses supplémentaires ou encore la suppression de la réforme relative aux redevances des agences de l'eau, notre groupe s'abstiendra sur cette première partie du projet de loi de finances pour 2024. Merci, cher collègue. Je passe enfin la parole à monsieur Kozik pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez cinq minutes, cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La première partie du budget que nous venons d'examiner s'inscrit dans un contexte de de contrainte budgétaire qui ne veut pas encore dire son nom. Il est clair que le retour à bas bruit des politiques austéritaires semble poindre alors même que se financer sur les marchés devient de plus en plus coûteux. Dans le même temps, la poussée de fièvre inflationniste qui frappe le pays n'en finit plus de ne pas finir. A cela s'ajoutent les diverses crises internationales qui s'amoncèlent au port de l'Europe et du Moyen-Orient, accentuant aussi la tension sur les marchés ce qui met notre économie à rude épreuve et va impacter durablement nos politiques publiques. Une fois le contexte posé, revenons au présent texte examiné. Cette première partie recette aura été largement en-deçà des besoins, alors même que la dette se creuse, que les besoins en services publics et que les financements de la transition écologique se font de plus en plus attendre. J'y reviendrai plus en détail. Néanmoins, je note que pour ne pas apporter de piste de financement nouvelle, vous avez fait le choix de mettre sous le boisseau des débats essentiels tels que la fiscalité du capital ou la contribution des plus aisés à l'effort collectif de redressement des comptes publics. Nous le regrettons, car vous n'avez, durant nos nombreuses heures de séance, eu de cesse de regarder ailleurs. Suppression de la flat tax, ISF vert, taxation des dividendes, tout a été rejeté en bloc. Nous nous félicitons que, durant cet examen, le gouvernement aura été battu à plusieurs reprises. Nous sommes, contre votre avis, parvenus à revenir sur le recentrage du préto 0, la baisse des moyens des chambres consulaires. Nous avons souhaité avancer sur un dispositif encadrant les rachats d'actions de manière plus efficiente. Le compromis est certes moins dix ans, mais il a le mérite de poser un premier jalon. Sur la fiscalité du capital, une fois n'est pas coutume, votre tropisme à aider ceux qui n'en ont pas besoin s'est encore exprimé. Vous avez réussi l'exploit de coaliser tous les bancs de cet hémicycle contre vos aberrantes, avantageuses mesures fiscales en faveur des fédérations sportives internationales. Mesures qui, je le rappelle, avaient été ajoutées à la USART à la défaveur de l'utilisation du 49.3. Preuve, s'il en fallait du manque de sérieux d'un tel dispositif, nos collègues de la majorité présidentielle n'ont pas participé au vote effectué à main levée. C'est dire le malaise qui entoure ce dispositif que vous ne manquerez pas de rétablir après votre 20ème 49.3. Je dois le dire, durant l'examen de cette partie recette, il y a eu beaucoup de grands absents. Tout d'abord, et alors que l'INSEE indique que 9 millions de Français se sont trouvés en situation de privation matérielle et sociale en 2022, l'USH a pour sa part estimé à 518 000 le nombre de nouveaux logements sociaux dont nous avons besoin chaque année. A l'instar du dernier quinquennat, le logement aura été, une fois de plus, le véritable angle mort de ce budget. Je me félicite néanmoins que notre amendement, revenant sur l'avantageuse niche fiscale Airbnb, ait pu trouver une majorité sur ces bancs. Enfin, comme je l'avais dit lors de l'ouverture des des débats, il est des absents qui se font remarquer. En l'espèce, celui du financement de la transition écologique. À ce titre, nous regrettons vivement que notre amendement visant à restaurer un ISF vert n'ait pas trouvé écho sur ces bancs. Nous regrettons également votre fu de toute conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Enfin, nous déplorons que les revendications des collectivités territoriales n'aient pas pu être suffisamment entendues. Alors que leur situation financière est extrêmement difficile, la droite sénatoriale et le gouvernement ont refusé de voter notre amendement visant à indexer la DGF sur l'inflation. Je note que la droite n'a de cesse de se présenter en centre de la défense des territoires, mais qu'elle n'a pas jugé opportun de voter un amendement qui aurait donné plus de moyens à nos collectivités locales afin de proposer des services publics au plus près des besoins. C'est aussi regrettable que la coïncophonie qui a entouré l'étude des LRR. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, cette première partie nous laisse un goût amer, un goût d'inachevé, en ce qu'elle ne nous permet pas de soutenir nos collectivités territoriales, de trouver les recettes fiscales nécessaires afin d'engager les moyens financiers pour la transition écologique, tout en préservant une certaine justice sociale. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous ne voterons contre ce volet recette du budget 2024. Merci, chers collègues. Les explications de vote ayant été données, je vais mettre au voie l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Au terme de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Nom de votant 345. Nom de suffrage exprimé 322 pour 219 contre 103. Le Sénat a adopté. La première partie du projet de loi de finances pour 2024 est adoptée. En conséquence, le Sénat peut commencer l'examen d'émissions de la seconde partie. M. le Ministre, vous voulez vous exprimer ? Vous avez la parole, M. le Ministre. Merci, M. le Président. Je vais vous dire peut-être quelques mots très très rapides parce qu'on aura passé quasiment 70 heures ensemble, si nos comptes sont bons. Et j'aime toujours voir le verre à moitié plein dans nos échanges parce que j'ai souvent dit défavorables et je pense que cette parabole du verre de vin ne vous déplaira pas. Non, moi je pense que quand même le Sénat, en votant cette première partie, on se retrouve sur quelques grandes priorités. Sur la transition écologique, sur la taxation des grandes infrastructures, sur les crédits d'impôt que nous avons, vous avez voté sur le bonus et le malus automobile. Sur le GNR, je trouve qu'on s'est retrouvés. On s'est retrouvés sur le soutien à l'activité économique. La baisse progressive de la CVAE a été votée ici, tout comme le crédit d'impôt industrie verte. Autant de dispositifs qui vont soutenir nos entreprises. Le troisième axe, qui est un axe fort de notre projet de loi de finances, que vous avez validé dans ces grandes lignes, l'impôt minimal sur les sociétés de 15%. l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, qui est une mesure attendue en termes de pouvoir d'achat, les mesures de lutte contre la fraude fiscale sur lesquelles nous nous sommes retrouvés. Tout en, je le dis, parce qu'il m'arrivait de plaisanter avec le rapporteur général sur le compteur et d'ailleurs sénatrice d'évoquer, sans trop dégrader la trajectoire. Il y a une petite amélioration en trempe-l'œil parce que vous avez voté une augmentation du prix de l'électricité de 20% en contrepartie d'un chèque qui arrivera en deuxième partie. Mais je suis satisfait que là, à ce stade, on maintient ce qui est notre objectif politique sur lequel on ne reviendra jamais, c'est le 4,4% de déficit. Pour l'instant, on est dans cette trajectoire-là. Alors naturellement, on a quelques divergences. Ça a été évoqué par le sénateur sur la suppression de la réforme des redevances de l'eau, qui sont la mise en œuvre du plan haut et qui décalerait cette réforme d'une année. Sur les collectivités territoriales, ça a été un peu houleux à un moment. Je réaffirme que vous avez été probablement trop loin dans le soutien aux collectivités territoriales. Et enfin sur le prix d'électricité, Le prix de l'électricité, le prix de l'électricité où on a un désaccord, on a pris l'engagement de ne pas augmenter le prix de l'électricité de plus de 10%, nous ne souhaitons pas aller au-delà, même s'il y a un mécanisme annoncé. J'ai pris des engagements ici pour continuer le travail avec vous sur un certain nombre de sujets, je pense à la TASCOM, je pense aux ESPIG en particulier, puis à la fiscalité du logement sur lequel il faudra quand même malgré tout y revenir. Et je voudrais terminer en remerciant naturellement le président. le rapporteur général, toutes celles et tous ceux qui sont restés très longtemps avec nous pendant ces discussions. Je voudrais avoir un mot aussi pour toutes les équipes du ministère de l'économie et des finances parce qu'on sait que le nombre d'amendements et les délais dans lesquels nous devons les examiner leur demande d'une grande mobilisation et associer aussi aussi mes remerciements aux équipes du rapporteur général très mobilisés dans cette période. Voilà et je vous dis pour ma part à bientôt parce que je vais passer le relais à mes collègues qui viendront défendre les crédits de la P2. Merci. Merci Merci Monsieur le Ministre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h pour l'examen de la mission sécurité du projet de loi de finances 2024. La séance est suspendue.